La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 14 février 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. Mes chers collègues, afin de permettre à ceux d'entre nous qui le souhaiteraient de se rendre au rassemblement contre l'antisémitisme qui se tiendra ce soir à Paris sur l'initiative de nombreux partis politiques, nous pourrions lever nos travaux à l'issue de notre séance de questions d'actualité au Gouvernement. Le débat sur les relations entre l'État et les sociétés autoroutières, demandé par le groupe Union Centriste, serait alors reporté à une date ultérieure fixée lors de la prochaine réunion de la conférence des présidents. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ! Nous sommes venus ici à Paris, bien déterminés à défendre et à obtenir ne serait-ce que des dispositions tendant à améliorer le fonctionnement de nos diverses institutions et à clarifier les compétences dûment réparties

Eh oui, mes chers collègues ! Les projets de loi que nous nous apprêtons à voter constituent une réelle avancée pour la Polynésie française. Il faut le souligner, ces deux textes ont été enrichis par l'adoption de nombreux amendements et ils sont le fruit de discussions intenses entre tous les niveaux de responsabilités, aussi bien en Polynésie qu'à Paris. La tâche a été rude, mais nous repartirons au avec le sentiment du travail bien accompli au titre de ce toilettage de la loi statutaire. La reconnaissance du fait nucléaire, inscrite dans la loi, est un grand pas de l'État, pour lequel nous n'avons pas ménagé nos efforts. Le fait nucléaire fait partie de notre histoire. Il constitue la pierre angulaire de l'accord de l'Élysée pour le développement de la Polynésie française au sein de la République, et il convenait de l'inscrire dans le marbre de notre loi statutaire. Notre économie insulaire a été profondément touchée, lors de l'installation du centre des expérimentations atomiques, puis lors de l'arrêt définitif des essais nucléaires, prononcé en 1996. Une reconversion s'est imposée, immédiatement engagée par le pays et fortement soutenue par l'État, en compensation de la baisse d'activités. Mais les impacts sanitaires, environnementaux et économiques se font toujours sentir. Cette reconnaissance qu'apporte le projet de loi organique est ainsi profondément symbolique et largement méritée, pour ne pas dire légitime, madame la ministre. Au-delà du fait nucléaire, le projet de loi organique comprend plusieurs dispositions permettant un fonctionnement plus efficient de nos institutions polynésiennes. Il assure non seulement davantage de stabilité à l'assemblée de la Polynésie française- l'erreur « matérielle » de dissolution de l'assemblée,

la parité sera garantie au sein du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Les modalités de gestion des membres de cette institution sont adaptées, le partage des compétences entre les communes et le pays est redéfini et renforcé.

l'outre-mer. Il assouplit le régime contentieux des lois de pays lorsque le Conseil d'État n'a pas statué dans un délai de trois mois. Ainsi, la loi sera promulguée en Polynésie sans plus attendre. Toutes ces nouvelles dispositions contribueront à un meilleur fonctionnement des institutions locales. Pour sa part, le projet de loi ordinaire nous permet notamment d'apporter enfin des réponses au grave problème de l'indivision successorale que nous connaissons en Polynésie. Les enjeux sont considérables pour un territoire comme le nôtre, et seuls des dispositifs spécifiques pouvaient y répondre. Nous nous réjouissons de leur mise en oeuvre prochaine au sein du tribunal foncier créé à Papeete. Par ailleurs, une adaptation de quelques articles du code général des collectivités territoriales, pour le compte de nos communes, s'avérait nécessaire, et le dispositif des crématoriums est enfin étendu à la Polynésie française. Nous pouvons nous féliciter de ce que ces deux projets de loi, dans leur ensemble, permettent que nos spécificités soient mieux que jamais prises en compte. Je rappelle que 16 000 kilomètres nous séparent de Paris là non pas des faveurs que nous demandons, mais bien des besoins que nous exprimons au titre du droit à la différenciation. La République française est riche de la diversité que recèle l'ensemble de ses territoires ultramarins. La zone Pacifique représente une des richesses maritimes de la France. Située aux antipodes de l'Europe, elle ne doit pas être négligée, d'autant qu'aujourd'hui l'axe indopacifique est largement convoité. Notre attachement à la République française n'en est que plus fort. En outre, la venue annoncée du Président de la République sur notre territoire est une occasion, pour la France, d'affirmer une véritable stratégie géopolitique et économique pour les décennies à venir. Pour finir, finir, je remercie de nouveau, en mon nom propre, mais aussi au nom du président Édouard Fritch, le président du Sénat, Gérard Larcher, mon président de groupe, Hervé Marseille, ainsi que que tous les autres présidents de groupe de leur soutien dans la préparation et l'examen de ces deux textes de loi. Nous vous remercions également, madame la ministre, de votre coopération et de votre action au service de la Polynésie française.

: servir l'intérêt général et contribuer au développement durable de la Polynésie française. Je ne doute pas du soutien que mes collègues, de toutes les travées, m'apporteront lors du vote de ces deux projets de loi essentiels au fonctionnement des institutions de notre si belle Polynésie française. ! La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, reconnaître la « dette nucléaire » de la France à l'égard de la Polynésie française, faciliter l'exercice de ses compétences par le pays, garantir la stabilité des institutions territoriales et faciliter le règlement des difficultés foncières polynésiennes tels sont les objectifs auxquels répondent le projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles. S'il est dépourvu de valeur normative, l'article 1 du projet de loi organique est hautement symbolique. La France a procédé à 193 essais nucléaires en Polynésie française entre 1966 et 1996, cette reconnaissance de la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire française est juste et nécessaire. Juste et nécessaire aussi est l'engagement de la République à en assumer les conséquences, qu'il s'agisse de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, de l'entretien et de la surveillance des sites d'expérimentation ou de la reconversion de l'économie polynésienne à la suite de la cessation des essais. Je me réjouis que, lors de ses travaux, la commission des lois ait adopté un amendement du Gouvernement tendant à ce que l'État informe, chaque année, l'assemblée de la Polynésie française des actions mises en oeuvre sur cette base. en oeuvre sur cette base. Le projet de loi organique vise également à faciliter l'exercice par la Polynésie française de ses compétences, en diversifiant les moyens dont elle dispose à cet effet, en précisant les attributions de ses institutions et en clarifiant les modalités de sa coopération avec l'État et avec les communes ou autres personnes publiques polynésiennes. polynésiennes. Les articles 12 et 13 du projet de loi organique visent, quant à eux, à garantir la stabilité des institutions polynésiennes. En effet, les dispositions actuelles du statut, très ambiguës, peuvent sembler imposer le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française dès lors que trois de ses membres démissionneraient simultanément. Aussi, je me félicite de ce que la commission des lois ait consolidé le dispositif proposé par le projet de loi organique. Désormais, les sièges devenus vacants pour quelque cause que ce soit le resteront jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée, sauf si leur nombre atteint le tiers de l'effectif légal de l'assemblée, auquel cas il y aurait lieu de renouveler cette dernière par anticipation.

d'autre part, elle a souhaité conserver la possibilité, pour les communes polynésiennes, de créer un syndicat mixte ouvert ne comprenant ni la Polynésie française ni l'un de ses établissements publics. Elle a également défini les dispositions applicables dans le cas où des communes ou groupements participeraient au capital de sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française ou ses établissements publics. Par ailleurs, la commission a introduit dans le projet de loi des dispositions visant à faciliter la sortie de l'indivision foncière en Polynésie française, pour mettre fin à des situations inextricables qui entravent l'exploitation des terrains. Enfin, elle a adopté quelques mesures d'ajustement visant notamment à autoriser les communes polynésiennes à créer et à gérer des crématoriums et des sites cinéraires ainsi qu'à moderniser le statut des 673 agents non fonctionnaires de l'administration. Avant de conclure, je souhaite, à cette tribune, saluer le travail du rapporteur, notre collègue Mathieu Darnaud. Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants n'a aucune réserve à émettre sur ces deux textes très attendus en Polynésie française. correspondent à un dialogue approfondi avec les élus polynésiens. Aussi, le groupe Les Indépendants les votera ! La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la République est non pas une administration hexagonale, mais une conception de la France qui traverse les siècles comme les océans.

Rapporteur de ces deux textes, j'ai pu observer que tous les acteurs concernés- exécutif et assemblée de la Polynésie, Gouvernement et élus locaux polynésiens -avaient à coeur de faire converger leurs vues, afin que la navette parlementaire soit aussi consensuelle que rapide. C'est dans cet esprit d'ouverture que les amendements adoptés en commission des lois, ou présentés par le Gouvernement, ont pu être acceptés par les différents interlocuteurs. Collectivement, grâce à cette concertation poussée, nous avons su élaborer un texte négocié, et ce sans avoir immolé les nécessaires réformes sur l'autel du compromis. Je tiens donc à souligner les avancées rendues ainsi possibles ; elles touchent notamment à trois domaines. de loi organique, du fait nucléaire, de la contribution de la Polynésie française à la dissuasion nucléaire. Cette dernière étant la pierre angulaire de notre système de défense, on mesure le rôle que ce territoire d'outre-mer a joué pour notre sécurité, mais aussi pour l'autorité de la voix de la France dans le monde. Il est juste de reconnaître cette contribution d'importance, de même qu'il est indispensable d'indemniser mieux et plus vite les victimes de nos campagnes d'essais nucléaires ; et c'est l'honneur d'un grand pays comme la France de considérer avec dignité ceux qui ont eu à subir les conséquences des essais dans leur chair. au travers de ces projets de loi, nous avons abordé les questions du règlement des difficultés foncières et des indivisions. Ces dernières sont particulièrement prégnantes dans nos collectivités d'outre-mer, et je tiens à à saluer le travail considérable accompli par la délégation sénatoriale aux outre-mer, que préside notre collègue Michel Magras. En s'appuyant sur les trois rapports qu'elle a publiés le Sénat a oeuvré pour sortir des situations inextricables créées par le phénomène d'indivision successorale, véritable obstacle à la construction et, donc, au développement de ces territoires. Troisièmement, l'exercice et la répartition des compétences, ainsi que le fonctionnement des diverses institutions polynésiennes dans le cadre du statut d'autonomie prévu par l'article 74 de notre Constitution, Cette autonomie est une nécessité : il ne s'agit pas moins que d'administrer un territoire dont les réalités sont celles d'un archipel constitué de 118 îles dispersées sur une superficie équivalant à celle de l'Europe-rien que L'exemple polynésien illustre combien, dans la gestion des compétences de nos collectivités, l'équité appelle non pas l'uniformité, mais l'imagination. On touche ici pleinement au principe de différenciation territoriale. Voilà pourquoi, désormais enrichis par le Sénat, ces textes vont, sans ébranler le statut général de la Polynésie, faciliter l'exercice des responsabilités dans ce territoire. Seront ainsi améliorés le fonctionnement des autorités administratives indépendantes, le régime juridique des sociétés publiques locales et et des sociétés d'économie mixte, avec chaque fois le même objectif : adapter les instruments aux spécificités locales. Le partage des compétences entre le pays, les communes de Polynésie et les diverses institutions présentes en Polynésie a également été clarifié, et les lois de pays adoptées par l'assemblée de la Polynésie seront plus facilement applicables. L'impact des décisions votées par cette assemblée en sort ainsi conforté, rendant l'action publique plus perceptible, au bénéfice de la vitalité démocratique. Quant aux institutions,

Enfin, le texte s'est enrichi de nombreuses avancées, parmi lesquelles le régime des syndicats mixtes, le recouvrement de l'impôt, l'encouragement à l'intercommunalité, ou encore la modernisation du statut des agents non fonctionnaires de l'administration. Toutes ces dispositions techniques permettront d'apporter de l'huile dans le meccano des diverses institutions polynésiennes. Gageons que ces dernières seront plus faciles à piloter, et que le service rendu à la population n'en sera que meilleur.

Ces deux projets de loi n'en constituent pas moins de réels progrès, de réelles avancées : c'est la raison pour laquelle les sénateurs du groupe Les Républicains les voteront avec confiance. Forte de cette évolution, la Polynésie sera mieux armée pour regarder l'avenir avec sérénité et répondre aux défis qui s'annoncent dans cette région du globe. C'est au coeur de l'océan Pacifique que se jouera demain une grande partie de l'avenir du monde ; la Polynésie sera alors, avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, en première ligne pour porter la voix de la France ! La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ces deux textes, attendus depuis plusieurs années par la Polynésie française, sont le fruit d'échanges anciens, nourris et riches, entre les élus polynésiens, le ministère des outre-mer et la commission des lois du Sénat, par la voix de son rapporteur. Ils sont la traduction législative de l'accord du 17 mars 2017, qu'ont signé François Hollande, alors Président de la République, et Édouard Fritch, président de la Polynésie française, et que le Président de la République actuel, Emmanuel Macron, a tenu à honorer. Nous sommes tous d'accord pour affirmer que le toilettage des textes statutaires et institutionnels polynésiens opéré par les deux projets de loi est indispensable au bon fonctionnement de ce pays d'outre-mer. nous l'avons indiqué au cours de la discussion générale : ces deux textes contiennent à la fois un symbole fort, répondant à une demande ancienne- la reconnaissance par l'État du fait nucléaire et de ses conséquences -, et de nombreuses dispositions techniques. Ils corrigent des dispositions du statut, telles que les conventions soumises à l'assemblée ou encore les délégations de signature, qui posaient des difficultés dans le fonctionnement des institutions polynésiennes. Ils clarifient également le partage des compétences entre l'État et le pays, en conférant à ce dernier la possibilité de créer des sociétés publiques locales, de participer à des syndicats mixtes ouverts, de constituer une autorité administrative indépendante de régulation dans un champ relevant de ses compétences et d'adhérer à un plus grand nombre d'organismes internationaux. Pour favoriser la création de communautés de communes et de syndicats mixtes en Polynésie française, le projet de loi ordinaire modifie des dispositions du code général des collectivités territoriales. Partant de bonnes intentions, un certain nombre d'amendements ont été déposés par nos collègues et rejetés par la Haute Assemblée. Il me semble primordial de faire confiance à la Polynésie française. Bien sûr ! Cette confiance aux territoires, nous l'appelons régulièrement de nos voeux dans cet hémicycle ; c'est justement en cela que les présents projets de loi sont intéressants, car ils répondent à cette volonté de prendre en compte la différenciation et le dialogue.

le rapporteur et moi-même étions les auteurs et que nous avions formulées à l'issue d'un déplacement très enrichissant dans le Pacifique. En séance, le Gouvernement a soutenu la demande forte des Polynésiens de pouvoir créer de nouvelles autorités administratives indépendantes. je vous sais femme de dialogue ; et je souhaite saluer le gage fort donné par le Gouvernement de sanctuariser la dotation globale d'autonomie en la retirant du budget du ministère des outre-mer et en la transformant, à l'instar de la en un prélèvement sur recettes dès 2020. Je l'indiquais lors de la discussion générale : il ne fait aucun doute que ces textes, marquant la volonté du Gouvernement d'entretenir une relation de confiance avec les autorités polynésiennes, sont porteurs d'avancées réelles pour nos compatriotes polynésiens. Voilà pourquoi, vous l'aurez compris, le groupe La République En Marche les soutiendra

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, répondant à une revendication exprimée de longue date par les Polynésiens, ces deux projets de loi renforcent le statut d'autonomie de la Polynésie en permettant un réajustement équilibré des compétences entre l'État et les institutions polynésiennes. Cette modernisation représente une avancée décisive, et nous ne pouvons que nous féliciter de ces mesures. Surtout, nous saluons le symbole fort de la reconnaissance par l'État français du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de la politique française de dissuasion nucléaire. Ces expérimentations nucléaires ont affecté l'environnement et la santé des Polynésiens pendant plus de trente ans. Ce lourd tribut a longtemps été minimisé par les politiques publiques ; la mesure déclarative dont il s'agit constitue donc un grand progrès. cette reconnaissance dénuée de réelle portée normative contraignante nous interpelle. Les réglementations en matière d'ouverture à l'indemnisation des personnes victimes des rayonnements nucléaires ne sont pas optimales ; en atteste notamment le fait que, entre 2010 et 2017, seules 42 indemnisations ont été obtenues pour 1 245 dossiers déposés. Pour 2018, le rapport de la commission de cadrage de la loi d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a abaissé le seuil d'exposition aux rayonnements en vigueur, qui constituait un frein dans le traitement des demandes, permettant ainsi d'accorder des indemnisations à 75 dossiers supplémentaires. Cette nouvelle mesure constitue un progrès, mais n'est, hélas, pas pleinement satisfaisante. Nous appelons donc de nos voeux la levée totale des obstacles majeurs aux demandes d'indemnisation. Les Polynésiens ont déjà trop attendu et doivent obtenir une juste réparation. règne également s'agissant de l'intervention de l'État pour assurer la dépollution des atolls affectés par les essais nucléaires, lesquels ont été profondément touchés par la pollution liée aux métaux lourds. Nous regrettons que le texte ne fasse pas mention d'un véritable investissement de l'État afin de réparer les nombreux préjudices écologiques subis dans les îles. les îles. Sur le plan environnemental, le texte présente une autre lacune : l'absence de normes protectrices de la biodiversité encadrant les activités d'exploration et d'exploitation minière des eaux intérieures polynésiennes.

Les explorations marines doivent se faire dans le strict respect de nos engagements internationaux. À l'article 9 de ce texte, lequel précise le cadre juridique de l'exploitation des terres rares, les mesures contraignantes de nos conventions internationales en la matière. La commission La commission a réalisé un important travail sur le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie, consacrant des avancées positives en matière de droit des successions. La Polynésie était en proie à d'importantes difficultés foncières, car des lacunes au niveau de l'état civil et du cadastre ne permettaient pas l'identification claire des ayants droit. Durant de nombreuses générations, ces difficultés se sont traduites par une absence de règlement des successions. Nous saluons donc les nouvelles dispositions, dérogatoires au droit commun, instaurent plus de souplesse dans les sorties d'indivision et protègent les conjoints survivants grâce à l'usufruit. Enfin, la Polynésie française dispose de nombreux atouts qui permettront son développement économique. L'adaptation du statut de la Polynésie a tenu compte des particularités de ce territoire, composé d'archipels très étendus : des autorités administratives indépendantes, des sociétés publiques ainsi que des syndicats mixtes

Le renforcement de l'intercommunalité voté dans le présent projet de loi permettra également de redynamiser le tissu économique local. Mes chers collègues, ce n'est franchement

faut imaginer 118 îles réparties sur un territoire plus grand que l'Europe, à 16 000 kilomètres de notre métropole,

! Il a fallu qu'à cette tribune Victor Hugo fît trois discours pour que, quelques années plus tard, il y eût cette amnistie pour la Commune de Paris. Je me permets de le dire, parce que ces événements sont importants dans notre histoire, mes chers collègues. Le texte dont nous parlons aujourd'hui, madame la ministre, est la traduction de l'accord signé le 17 mars 2017 par François Hollande et Édouard Fritch, président de la Polynésie française. Le Président de la République avait alors déclaré : « C'est un accord d'abord politique, qui met la Polynésie pleinement dans la République. Cette place ne doit jamais être remise en cause. » Madame la ministre, je vous ai déjà dit que vous incarniez la continuité et vous êtes sans doute satisfaite que le président Emmanuel Macron

Tout s'est donc passé dans de bonnes conditions. L'accord que ce texte va inscrire dans la loi la loi est important pour la Polynésie française, non seulement en matière institutionnelle, mais également pour des raisons de fond qui tiennent à son nécessaire développement économique. La Polynésie

mais aussi avec le souci de faire vivre dans les meilleures conditions possible l'ensemble des Polynésiens grâce à un développement économique maîtrisé. Se posent aussi le problème de la continuité territoriale, que vous connaissez bien, la question du désenclavement, à la fois aérien et numérique, ainsi que celle du développement touristique, qui permette de faire connaître en profondeur la richesse de la Polynésie et tout ce qu'elle peut apporter en termes non seulement de soleil et de mer, ce qui n'est pas négligeable, mais aussi d'humanisme, de philosophie et de rapport avec la nature.

que les sommes sur lesquelles vous vous êtes engagée, madame la ministre, soient bien inscrites dans les lois de finances, de manière que cette indemnisation aille enfin à son terme dans des délais rapprochés. Il y a une injustice à l'égard des victimes : vous vous êtes engagée à la réparer ; il faut le faire dans des délais très rapprochés. Je terminerai en rappelant que nous avons marqué quelques différences, quelques nuances, s'agissant, tout d'abord, des autorités administratives indépendantes.

De même, nous pensons que les sociétés publiques locales peuvent apporter une souplesse nécessaire, à condition que leur objet soit public. Nous l'avons dit, nous y tenons. J'ai remarqué que vous aviez appelé à la sagesse sur l'amendement que nous avions déposé nous avions déposé à ce sujet ; ce n'était pas anodin de votre part. Enfin, s'agissant du statut des personnels, nous sommes très attachés à l'égalité et il nous semble que la référence au statut des personnels des assemblées parlementaires n'était pas pertinente puisqu'il s'agit, après tout, de collectivités locales. Moyennant quoi nous considérons que ce texte est un progrès pour la Polynésie française, pour tous ses habitants et toutes ses habitantes. C'est pourquoi notre groupe

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au moment de dresser le bilan de l'examen de ces deux textes, je tenais tout d'abord à souligner la qualité de nos échanges. Je félicite notre rapporteur Mathieu Darnaud, qui n'a pas ménagé ses efforts pour tenir compte des opinions exprimées par les différents groupes, en essayant toujours d'apporter des réponses aux problèmes soulevés, dans le souci permanent de parvenir au texte le plus consensuel possible. Mes félicitations s'adressent également à vous, madame la ministre, d'abord pour avoir déposé ces deux projets de loi attendus de longue date. Vous avez su faire preuve d'ouverture d'esprit durant nos débats, même si, en Ultramarine que vous êtes, vous avez des convictions fortes et vous les exprimez Mes chers collègues, au cours des discussions, le groupe du RDSE a souhaité attirer votre attention sur deux points, sur lesquels j'aimerais revenir brièvement. brièvement. En notre qualité de législateur et parce que nous légiférons pour l'avenir, nous avons tout d'abord jugé indispensable que soient questionnées les dispositions relatives aux autorités administratives indépendantes, objets de nombreux rapports au cours des dernières années

la prolifération de ces autorités [ ...] contribue de plus en plus fortement à l'illisibilité et au dysfonctionnement du système institutionnel, alors même que la volonté de simplification administrative doit constituer une ardente obligation afin de redonner tout son sens et son efficacité à l'action publique ». C'est donc uniquement par cohérence avec ces recommandations que nous avions déposé un amendement tendant à supprimer l'article 4, et non pour nous opposer d'une quelconque manière à la volonté des autorités polynésiennes. Suivant la même idée, il nous a semblé cohérent de rappeler les dispositions contenues dans la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales, adoptée en 2010, qui fixaient comme exigence exigence le maintien d'une présence obligatoire de deux actionnaires au minimum, alors que l'article 5 du présent texte offre la possibilité d'un actionnaire unique. Notre groupe a, lui aussi, su faire preuve de sagesse : après avoir écouté avec attention les observations et les arguments avancés à la fois par le rapporteur et par vous-même, madame la ministre, pointant les spécificités locales, nous avons fait le choix de retirer nos deux amendements. C'est, je le crois, la grande force de notre assemblée que d'arriver très régulièrement à dépasser les postures et les clivages partisans pour écouter, échanger, débattre et parvenir, le plus souvent, au consensus.

Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. » Aussi, je tiens à témoigner au peuple polynésien même si des dispositifs viendront apporter un dédommagement aux victimes, nous avons conscience que les blessures physiques et morales ne pourront jamais se refermer complètement. Aucune compensation financière ne saurait être juste ou équitable, tout simplement parce que la vie n'a pas de prix. Nous saluons, néanmoins, les avancées qui permettront d'améliorer ces dédommagements. Je forme le voeu que ces deux textes permettent aux autorités polynésiennes de disposer des outils nécessaires à leur développement institutionnel et économique,

Je sais que nos amis polynésiens auraient souhaité aller encore plus loin, mais il faut laisser du temps au temps. Ces projets de loi organique et ordinaire, qui viennent compléter la loi de 2004, sont voués, eux-mêmes, à être enrichis à l'avenir.

Le territoire de Saint-Martin, après dix ans d'existence, a suffisamment de recul pour évaluer les limites de son statut actuel.

Madame la présidente, madame la ministre, j'ai pu constater qu'il y avait un large consensus sur ce projet de loi organique. Cela prouve que le texte répond à un besoin et qu'une

Il est des domaines où, manifestement, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas allé trop loin. Par exemple, lorsqu'avaient été examinés, il y a quelques mois, les textes sur la Nouvelle-Calédonie, j'avais exprimé mon opposition radicale au fait qu'il y ait deux sortes

territoriales d'outre-mer. Mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi organique

Je remercie nos collègues Éric Bocquet, Françoise Gatel et Michel Raison, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je déclare le scrutin ouvert pour une demi-heure et je suspends la séance jusqu'à seize heure à laquelle je proclamerai le résultat. À l'issue, nous procéderons, dans l'hémicycle, au vote sur l'ensemble du projet de loi ordinaire. Je compte sur votre présence tout à l'heure. La séance est suspendue.

Le Sénat a adopté le projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'unanimité exprimée démontre que les deux textes sont de grande qualité : le travail a été conduit dans

L'État prend ici, vous le savez, des engagements importants concernant, tout d'abord, le dispositif d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, profondément rénové en 2018,

Les élus polynésiens, les acteurs économiques et les professionnels du droit considèrent à juste raison et unanimement que le droit applicable est aujourd'hui d'une complexité énorme et souvent Comme vous l'avez souhaité, monsieur le rapporteur, l'État lancera une mission sur la lisibilité du droit en Polynésie.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes très chers collègues, ce qui fait l'actualité, hélas, ce sont des actes d'une ignominie telle qu'ils remettent en cause la nature même de notre pacte républicain. Ce sont le lâche assassinat de Mireille Knoll, la mémoire d'Ilan Halimi et de Simone Veil outrageusement bafouée, l'agression d'Alain Finkielkraut, la profanation d'un cimetière juif aujourd'hui même en Alsace, que nous découvrons avec horreur. Parfois, sous couvert d'antisionisme, les comportements les plus abjects sont permis. Mais gardons-nous, monsieur le Premier ministre, de la tentation d'un nouveau texte de loi élaboré dans l'émotion. Notre arsenal législatif ne nous permet-il pas, déjà, de répondre avec la plus grande des fermetés ?

de plus en plus fragmentée, de plus en plus vulnérable à la manipulation de l'information et des faits historiques ainsi qu'à la propagation d'idéologies haineuses, à l'opposé de nos valeurs républicaines. Il est, à cet égard, nécessaire de réguler internet et les plateformes, qui permettent tous les débordements. Le Sénat a formulé des propositions très fortes à cet égard. Mais aussi et surtout, il convient de ne pas laisser s'installer l'idée que l'antisémitisme serait une opinion comme une autre. Cela passe d'abord, monsieur le Premier ministre, par des précisions, qui doivent être apportées à la lettre adressée par M. le ministre de l'éducation nationale, le 31 août 2018, aux enseignants, où il est question du respect d'autrui, de la transmission de savoirs fondamentaux et de l'éducation aux valeurs de la République. Le Sénat examinera prochainement le projet de loi pour une école de la confiance. C'est un véhicule idéal pour permettre aussi de rappeler l'importance et la réalité des faits historiques ainsi que l'importance d'une éducation aux médias et au numérique, encore largement insuffisante aujourd'hui. Tout nous oblige à un véritable sursaut républicain, mes chers collègues. À l'appel des formations politiques, le grand rassemblement de ce soir à Paris et dans la France entière est très important. Mais, au-delà, monsieur le Premier ministre, quelles mesures vont être prises pour reconstruire ensemble,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Morin-Desailly, vous avez commencé votre question en rappelant une série de faits, d'actes ou de propos antisémites. Ces faits, nous les connaissons, certains ont été rendus visibles

Vous avez indiqué que nous devions dénoncer ces faits et vous avez rappelé la marche ou, plus exactement, le rassemblement qui sera organisé ce soir à à Paris et dans de très nombreuses villes françaises. Ces rassemblements sont nécessaires ; ils sont utiles pour que nous puissions tous ensemble, sans exclusive, dire que ces faits sont inacceptables. Mais ils ne sont pas suffisants, et nous en avons parfaitement conscience.

nous ne devons pas nous contenter d'une dénonciation morale : nous devons la faire, mais nous ne devons pas nous en contenter. Évidemment, le champ de l'action est considérable. Je pense d'abord et avant tout à l'éducation et au soutien aux enseignants quand ils transmettent l'histoire, les faits, qu'ils sont confrontés à des propos ou à des actes antisémites ; je pense également à la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, qui concourent à réprimer ou à prévenir ces atteintes.

Je vous rejoins volontiers sur ce sujet, mais il ne faut pas non plus renoncer à légiférer lorsque cela est nécessaire. Or il y a au moins un champ- il en existe peut-être d'autres -où cela est parfaitement nécessaire, c'est celui des réseaux sociaux et d'internet,

écrivent, promeuvent des propos parfaitement antisémites et parfaitement inacceptables. Cette impunité ne peut pas prévaloir. Nous savons que le droit national- d'ailleurs, à bien des égards, pour le droit communautaire -n'est pas à ce jour adapté à la sévérité de la réponse que nous sommes en droit d'attendre. C'est la raison pour laquelle, à la suite d'un rapport qui a été préparé notamment par Mme la députée Avia, nous voulons compléter notre droit national et militer pour compléter le droit communautaire en en modifiant le statut de ceux qui gèrent des réseaux sociaux, en vue d'invoquer leurs responsabilités s'ils ne font pas ce qui est nécessaire pour retirer les publications sur ces réseaux sociaux, voire

en vaut la peine. Je crois profondément, madame la sénatrice, que nous devons légiférer : il ne serait pas acceptable qu'en matière d'antisémitisme nous donnions le sentiment que l'impunité pourrait prévaloir.

Je souhaite que, systématiquement, les affaires d'antisémitisme donnent lieu à des poursuites et je souhaite également que, systématiquement, elles donnent lieu à des sanctions sévères.

Il est question d'un rapport du préfet, de rencontres diverses ; bref, chacun y va de la sienne. Pour être synthétique sans être réducteur, le problème peut se résumer en quelques grands points. point, la fusion- faute d'un mot meilleur -entre métropole et département, en se souvenant aussi que le social constitue la plus grande partie du budget de fonctionnement et qu'il s'agit là d'une culture tout à fait à part. point, la question des vingt-neuf communes du nord du département, dont certaines sont regroupées autour d'un projet commun qui se voudrait expérimental ; je parle de la création d'une collectivité territoriale à statut particulier. point, le destin de deux communes hors département des Bouches-du-Rhône, Saint-Zacharie, dans le Var, et surtout Pertuis, dont le retour vers son département d'origine, le Vaucluse, ne fait pas l'unanimité. Capitale du nord du Lubéron, il est vrai que Pertuis est davantage tournée vers Aix, y compris pour ce qui

en rappelant que Marseille est une ville pauvre. Certes, il faut l'aider, mais ce n'est pas en appauvrissant les autres communes, dont les budgets sont déjà très fragiles, en touchant en particulier à leur attribution de compensation, que nous parviendrons à donner à Marseille son statut de capitale de métropole. Madame la ministre, quand y verrons-nous plus clair sur chacun de ces points ?

mais la ville de Marseille a également besoin de se renforcer. Reconnaissons-le, par ailleurs, Aix-Marseille est une réalité géographique et économique, qui couvre la quasi-intégralité du département des Bouches-du-Rhône. La métropole est, me semble-t-il, une chance pour les territoires et non pas une menace ; elle est le moteur d'une alliance des territoires et elle aussi une chance pour la ville de Marseille. Le Premier ministre a chargé le préfet de région, le préfet des Bouches-du-Rhône, M. Pierre Dartout, de mener une concertation afin d'étudier l'opportunité, les conditions et les modalités d'une fusion entre l'actuelle métropole et le département des Bouches-du-Rhône. Ce rapport sera rendu très prochainement et il éclairera le Gouvernement sur les points que vous avez soulevés : le périmètre de la métropole, la bonne répartition des compétences entre la métropole et les communes, ainsi que les moyens financiers bien sûr bien sûr et les questions électorales, sans oublier les territoires que vous avez cités au nord de la métropole. Ce sont autant de questions importantes parce que l'enjeu est de taille permettre à Marseille, à cette très grande ville française, à cette métropole méditerranéenne, de répondre aux défis du présent et de l'avenir pour tous les citoyens des Bouches-du-Rhône.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, de la démocratie représentative ? Devant le discours ambiant, nous ne pouvons masquer notre inquiétude pour celle que Pierre Rosanvallon qualifie de « seul horizon reconnu du bien politique ». Si certaines musiques comme la réduction du nombre de parlementaires ou d'élus locaux sont agréables à l'oreille de beaucoup de nos compatriotes, elles peuvent également se révéler pernicieuses. Le 14 février dernier marquait le cinquième anniversaire de la promulgation de la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat de député ou de sénateur. Au sein du Gouvernement et de la majorité, avec le recul, on s'interroge : le débat démocratique souffrirait-t-il désormais d'une forme de déconnexion de la représentation nationale ? En effet, ce qui était volontiers présenté comme un privilège était aussi souvent la garantie d'une politique ancrée dans la proximité, et ce jusqu'au sein du Parlement. Mais on estimait qu'une mesure aussi « populaire » devait être prise pour oeuvrer à la réconciliation des Français et de leurs représentants nationaux. Effectivement,

sur une réduction du nombre de parlementaires et d'élus locaux intervenue sous cette législature, quand les députés seront devenus invisibles au sein de circonscriptions de 200 000 habitants, quand près de la moitié de nos départements ne compteront plus qu'un sénateur ? Et d'une régionalisation de nos circonscriptions, qui conduirait un sénateur à sillonner un territoire allant d'Aurillac à Annecy ou de Bayonne à Poitiers, comme le souhaitent certains députés de la majorité

Monsieur le Premier ministre, alors que vous entendez faire évoluer nos institutions, saurez-vous conduire votre réforme tout en gardant à l'esprit que la légitimité du politique

garantit à tous, sans condition, « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » À défaut de respecter l'héritage de la Résistance, il conviendrait, au moins, de respecter la Constitution ! Vous parlez d'allocations

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour le groupe socialiste et républicain.

Sale juif, tu vas mourir » : voilà ce qu'il est encore possible d'entendre de nos jours, un samedi après-midi, au détour d'une rue de Paris, si, comme Alain Finkielkraut, on croise une délégation de « gilets jaunes », amalgame d'une ultra-gauche ou d'une droite fascisante et d'un islamisme radicalisé. Ce que nous vivons dans les rues de Paris, nous le retrouvons de manière décuplée sur internet, où l'antisémitisme côtoie le sexisme le plus primaire dans la plus grande impunité, comme l'affaire de la « ligue du LOL » l'a honteusement montré. Les lois existantes se révèlent insuffisantes. Il faut réformer, se donner les moyens d'agir contre la haine. Tout est prêt. Le rapport du 20 septembre 2018 visant à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur internet contient des propositions importantes, que nous devons adopter et appliquer au plus vite obliger les plateformes à retirer dans un délai de vingt-quatre heures tout contenu manifestement illégal ; fournir l'identité des auteurs ; multiplier par 100 le montant des amendes pour les moteurs de recherche et les réseaux sociaux qui manquent à leurs obligations

il faut légiférer au plus vite. Nos voisins Allemands ont récemment pris des mesures fortes, comme la nomination de chargés de mission contre l'antisémitisme, suivis en cela par la Commission européenne,

L'antisémitisme menace chaque jour davantage de personnes. Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, les discours haineux, le harcèlement, le sexisme prospèrent sur les réseaux sociaux. Nous attendons, de manière urgente, des actes forts de la part de l'État, pour mettre hors d'état de nuire toute personne qui répandrait la haine sur internet comme sur le sol de notre République. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour le groupe Les Républicains. « Il faut

des transports. Nous examinerons cette semaine en séance publique la proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires. Vous le savez, madame la ministre, les transports sont parmi les premiers facteurs de désenclavement d'un territoire.

Dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes conseille à l'État d'abandonner son rôle d'autorité organisatrice pour les trains d'équilibre du territoire, les TET, en raison de la faiblesse de ses moyens et des difficultés qu'il rencontre pour établir une relation contractuelle équilibrée avec la SNCF. Parmi les options envisagées figurent le transfert total de la compétence aux régions et le déconventionnement. Madame la ministre, vous l'avez vous-même rappelé, l'investissement de l'État dans le transport ferroviaire doit aujourd'hui répondre à une exigence de justice territoriale. années de financement des lignes à grande vitesse ont mis en péril l'avenir des trains d'équilibre du territoire. Parmi ces lignes structurantes, la ligne Paris-Clermont-Ferrand fait l'objet de toutes les attentions, en raison de son caractère stratégique et de l'engagement des élus, des acteurs économiques et des usagers. Le projet de loi d'orientation des mobilités, qui sera examiné au Sénat le mois prochain, prévoit de provisionner 760 millions d'euros pour la régénération de son infrastructure, deuxième volet d'un vaste programme de modernisation. Si nous nous réjouissons bien sûr de l'investissement de l'État sur cette ligne, nous nous interrogeons sur ses intentions à plus long terme, d'une part en raison du récent rapport de la Cour des comptes, d'autre part du fait de l'absence, dans le projet de loi d'orientation des mobilités, d'un engagement sur le financement du troisième volet de ce programme de modernisation, qui n'y est qu'évoqué. Madame la ministre, Madame la ministre, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour préserver, à plus long terme, ces lignes structurantes des trains d'équilibre du territoire ? La parole

Je serai claire, monsieur le sénateur : les lignes Intercités répondent à un objectif essentiel d'aménagement du territoire et je sais que les Français y sont très attachés. attachés. Ces lignes coûtent, effectivement, mais nous l'assumons totalement. La politique d'aménagement du territoire ne peut pas être traitée au travers d'une approche uniquement comptable.

Au contraire, le Gouvernement s'est engagé dans une modernisation sans précédent des trains d'équilibre des territoires. Ainsi, pour la ligne Paris-Clermont-Ferrand, le renouvellement des vingt-huit rames et la modernisation de l'infrastructure sont inscrits dans le projet de loi d'orientation des mobilités, qui sera débattu prochainement au Sénat. 700 millions d'euros est dédiée au renouvellement des trains et, par ailleurs, la réforme ferroviaire a permis de sécuriser les investissements de SNCF Réseau à hauteur de 3,6 milliards d'euros par an pendant dix ans. Ainsi, d'ici à 2025, la ligne Paris-Clermont-Ferrand sera équipée de trains neufs et aura été remise à niveau et modernisée. Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement se mobilise et s'engage en faveur de nos territoires, notamment en modernisant des lignes qui ont été trop

pour le groupe Les Républicains. Le Gouvernement a engagé de nombreuses réformes dans le domaine du handicap, mais beaucoup d'inquiétudes subsistent chez les acteurs et les familles. Six mois se sont écoulés depuis la promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont l'ambition était, notamment, de garantir un parcours professionnel plus fluide aux personnes handicapées.

Par ailleurs, madame la secrétaire d'État, pour qu'une personne handicapée puisse un jour espérer intégrer le milieu du travail ordinaire, ne pensez-vous pas que la priorité doit être d'investir dans sa formation dès les premières années ?

Qu'en est-il de la durée du contrat de travail, du niveau de rémunération, des formations- qui demeurent lacunaires -et des différences de traitement entre le public et le privé ? Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps

c'est le délai nécessaire à la préparation des textes d'application, bien sûr, mais aussi des outils nécessaires pour l'intégration dans la déclaration sociale nominative, la DSN, et des nouveaux services pour les employeurs et les personnes. Les concertations sont également engagées pour définir les nouvelles modalités de valorisation de la sous-traitance auprès du secteur du travail protégé et adapté. L'intention du Gouvernement est très claire est de continuer à valoriser le recours aux ÉSAT et aux entreprises adaptées, qui jouent un rôle majeur dans les parcours d'emploi de 150 000 travailleurs handicapés. La méthode repose sur le partenariat, que nous avons entendu renforcer au travers de l'engagement conclu le 12 juillet dernier avec l'Union nationale des Il va permettre la création de 40 000 emplois dans les entreprises adaptées d'ici à 2022, avec un soutien public porté à 500 millions d'euros. Voilà du concret ! Du concret, c'est aussi ce que nous apportons aux accompagnants des élèves en situation de handicap. Nous les avons pleinement associés à la concertation sur l'école

source de trop nombreuses ruptures pour les élèves et les accompagnants. Oui, plus d'accompagnants, monsieur le sénateur, et seulement des AESH recrutés sur de vrais emplois publics, des emplois « en dur » d'une durée minimale de trois ans renouvelable une fois : c'est le droit commun. C'est ensuite une vraie formation, des accompagnants comme des enseignants, ainsi que le prévoient les dispositions du projet de loi pour une école de la confiance, que vous serez bientôt amenés à examiner, mesdames, messieurs les sénateurs. Comme nous l'avions annoncé avec Jean-Michel Blanquer, la première lecture a permis d'enrichir un chapitre complet dédié au renforcement de l'école inclusive. Je sais pouvoir compter sur votre action pour continuer de progresser.

Républicains. Sous le quinquennat précédent, le pouvoir d'achat des familles s'est considérablement érodé, avec l'abaissement du plafond du quotient familial, la suppression de l'universalité des allocations familiales, l'abaissement des seuils de ressources pour bénéficier de la prestation d'accueil Le résultat ne s'est pas fait attendre : le taux de natalité a baissé pour la quatrième année consécutive. La garde de l'enfant de zéro à trois ans est une source de préoccupation. Le Président de la République annonçait récemment la création de nombreuses places de crèche. Si je loue la volonté exprimée, je suis très réservée sur les conditions d'application les municipalités toucheraient une subvention annuelle de 2 000 euros par place de crèche créée à la condition que les revenus des familles bénéficiaires ne dépassent pas 25 000 euros avec un enfant, 30 000 euros avec deux enfants. Le taux global d'accueil des enfants de moins de trois ans est le plus faible dans les zones où le marché de l'immobilier est tendu. Dans ces territoires, avec 2 500 euros par mois pour élever deux enfants et payer un loyer, vous êtes loin d'être riches ! Dit autrement, ce gouvernement propose aux mairies de créer des

pis, elle risque d'en supprimer, le reste à charge pour les communes ne cessant de s'accroître. Monsieur le secrétaire d'État, quand la France aura-t-elle un gouvernement qui prendra à bras-le-corps la politique familiale, pour la défendre et l'unifier ?

favorisant la mixité sociale dans les modes d'accueil du jeune enfant. Permettez-moi de revenir sur un certain nombre de ces dispositions, que nous assumons. Tout d'abord, le bonus « mixité sociale » et le bonus « territoire » du plan Pauvreté encouragent les gestionnaires et les villes à accueillir des enfants défavorisés, en compensant

L'attribution des places de crèche doit également être plus transparente. C'est sur ce point que je souhaiterais insister aujourd'hui devant vous. Je salue à cette occasion Élisabeth Laithier, chargée du dossier « petite enfance » au sein de l'Association

de François Baroin. La situation actuelle est insatisfaisante. L'insuffisance de l'offre d'accueil et la surreprésentation des enfants des ménages les plus aisés dans les modes d'accueil collectif alimentent un sentiment d'injustice sociale. En effet, vous le savez, seuls 5 % des enfants de moins de trois ans des 20 % de ménages les plus pauvres sont accueillis en crèche, contre 22 % des enfants des parents les plus aisés. La mission Laithier propose de mettre en place une grille d'attribution en sélectionnant des critères pertinents parmi un large socle existant, en fonction des spécificités de chaque territoire. Ce vade-mecum décrit les différents systèmes utilisés, tels que la priorisation, la bonification ou la pondération. Cette grille pourra être adaptée en fonction du suivi. C'est cette transparence et cette diversité dans l'offre d'accueil qui nous permettront d'assurer une meilleure coordination des acteurs et une meilleure harmonisation des pratiques entre les territoires. La parole

vient de s'achever à l'Assemblée nationale, je souhaite vous interpeller sur la situation des trente-deux écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les ÉSPÉ, qui forment aux métiers du professorat, de l'éducation et de la formation. Ces établissements sont également des composantes spécifiques, intégrées aux universités, que nous avions créés

vise, en effet, à les transformer en instituts, ce qui suscite des interrogations sur l'intention sous-tendant ce glissement de terminologie. Cette modification pourrait porter atteinte à la lisibilité de la formation des enseignants et des

pour réaliser de substantielles économies, ne serait-il pas opportun, en l'occurrence, d'appliquer la même règle à tous les niveaux de l'État ? Enfin, la concertation semble avoir été absente de l'élaboration de cette réforme. Les personnels expriment leur attente d'informations, d'autant que la mise en oeuvre est prévue pour la rentrée de septembre. Il est évidemment indispensable d'associer les enseignants aux évolutions, car eux aussi savent ce qui fonctionne ou pas. Alors que le mot « débat » fleurit sur toutes les lèvres, n'aurait-il pas été opportun de l'organiser en amont, avec tous les acteurs du monde éducatif ?

Nous aurons demain matin une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales pour évoquer cette réforme. Il est évidemment indispensable que, pour préparer cette nouvelle professionnalisation, et notamment une entrée accompagnée dans le métier,

Je vous remercie, madame la ministre, mais vous dites vous-même que vous continuez à travailler et à réfléchir : ce n'est pas rassurant pour la rentrée 2019 ... Je note en outre que vous n'avez pas répondu à la première question que je vous ai posée.

Lors d'une rencontre dans le Finistère, le Premier ministre a évoqué ses convictions personnelles concernant la mise en place de contreparties aux aides sociales. J'avoue avoir été extrêmement intéressé par sa démarche, car il s'agit d'un véritable projet de société, qui dépasse les clivages politiques habituels. Mais ce peut être un projet explosif s'il est mal compris ou mal construit Il s'agit non pas d'être punitif ou stigmatisant, mais d'inciter à réintégrer le monde du travail et d'assurer à la société le juste retour d'une solidarité nécessaire.

du parcours d'insertion des personnes. Le problème, nous le savons, est qu'aujourd'hui plus de 50 % des allocataires du RSA ne se voient proposer aucun contrat

Le bénéficiaire d'un contrat devra s'engager à suivre des formations, à accomplir certaines démarches ou à faire certaines activités pour favoriser sa réinsertion, dans le cadre des entreprises d'insertion vers l'emploi. Telle est l'idée qui sera soumise à consultation du grand public.